à l'occasion de chacun des débats que nous avons eus à ce sujet, que ce soit en PLFSS ou lors des différents PLFR, autant d'occasions de remettre l'ouvrage sur le métier ! Nous tenons à cet alignement et à cette convergence, tout en précisant qu'une qu'une fois cette convergence actée le régime de fiscalité sur les boissons visées par l'amendement restera un régime relativement plus favorable. La parole est à Mme Catherine Conconne, pour explication de vote.

12 % seulement de la production de rhum est consommée à la Martinique. Notre jeunesse et les locaux consomment davantage de bière importée, de cognac, de champagne non fabriqués chez nous et plus faiblement taxés. Imposer à cette filière, au potentiel de développement extraordinaire, un bâton supplémentaire dans ses moulins de broyage a été vécu comme une véritable injustice. injustice. Hélas ! chez nous, on a pris l'habitude et on s'est plié au rôle facile de financer l'inactivité, avec un RSA qui explose des chômeurs dont le nombre n'arrête pas d'augmenter. Mme la présidente du conseil départemental de Guadeloupe a souligné hier que plus de 1 000 Guadeloupéens supplémentaires étaient demandeurs du RSA depuis la crise du covid.

L'exonération de charges patronales pour les salariés de ces filières agricoles en grande difficulté a déjà fait l'objet de mesures adoptées à l'Assemblée nationale dans le projet de loi de finances (PLF) pour 2021. Il s'agit dans cet amendement de rendre accessible aux travailleurs non salariés agricoles une exonération de charges, car aucun dispositif n'a été prévu à leur égard alors même qu'ils subissent de plein fouet cette crise sanitaire qui affecte durablement leur activité. L'annonce d'un nouveau reconfinement, le 30 octobre dernier, va venir aggraver encore une situation déjà fortement dégradée et qui menace la survie de nombreuses exploitations ayant enregistré des pertes massives pendant la crise. Alors que les prix payés à la suite de l'effondrement du marché ne couvrent ne couvrent pas les coûts de production, que les reports de charges obtenus au printemps ainsi que les prêts garantis par l'État (PGE) souscrits vont devoir commencer à être remboursés sans réelle perspective de reprise dans les mois à venir, de nombreux exploitants vont verser dans la précarité. C'est pourquoi, afin de soutenir les petites entreprises agricoles pour lesquelles les cotisations sociales représentent une charge non négligeable, il convient d'attribuer cette exonération aux non-salariés de ces secteurs, en fonction des pertes subies au cours de l'année 2020. Elle permettra un réel allégement de leurs charges, en les exonérant de cotisations sociales pour 2020.

les non-salariés agricoles, c'est-à-dire les exploitants eux-mêmes, car beaucoup de petites entreprises viticoles n'ont pas forcément de salariés. Ces exploitations viticoles sont pourvoyeuses de centaines de milliers d'emplois non délocalisables sur l'ensemble de nos territoires, au travers de leurs activités saisonnières. Elles ont été terriblement impactées par la crise sanitaire, mais également économique. La consommation de vin associée aux événements festifs a fortement baissé, les salons sont annulés les uns après les autres, les exportations, notamment aux États-Unis, ont considérablement ralenti, les cafés, hôtels, restaurants sont fermés.

peut bénéficier. La viticulture est un ambassadeur de la France à l'international, un emblème de la gastronomie et de l'art de vivre à la française, qui est en train de se perdre. Elle est le deuxième contributeur positif de notre balance commerciale. une richesse, un patrimoine, une culture qu'il est essentiel de préserver. C'est la raison pour laquelle nous vous proposons une telle adaptation, en complément de l'article 13. L'amendement

Cet amendement a pour objet de défendre la filière viticole, qui a subi de plein fouet la crise économique liée à la lutte contre le coronavirus. Depuis plus d'un an, elle est en proie à un contexte économique difficile, que ce soit du fait du conflit entre l'Europe et les États-Unis sur l'aéronautique, dont la filière est une victime collatérale- les vins français sont taxés à 25 % depuis octobre 2019 à leur entrée sur le sol américain, qui est notre premier marché à l'export -, de l'enchaînement des difficultés à l'export- Chine, Royaume-Uni -ou encore de la crise sanitaire planétaire. Sur le premier semestre 2020, le secteur accuse des pertes de plusieurs milliards d'euros. Or, à l'inverse de nombreux secteurs économiques, les entreprises viticoles de la production n'ont pas eu recours dans leur très grande majorité au chômage partiel et ont continué à rémunérer leurs salariés pour assurer l'entretien de la vigne, en prévision de la récolte à venir. Le reconfinement en vigueur depuis le 30 octobre dernier va venir aggraver une situation déjà fort dégradée pour la fin de l'année 2020 ainsi que pour 2021 : pas de reprise du tourisme, notamment des visiteurs internationaux ; fermeture des bars et des restaurants ; annulation des grands salons professionnels et grand public ; reprise ; reprise en demi-teinte de l'export du fait de la situation sanitaire préoccupante dans de nombreux pays. C'est pourquoi, afin d'aider les petites entreprises pour lesquelles les cotisations sociales représentent une charge non négligeable, un soutien doit être mis en place en ce qui concerne les charges sociales des exploitants en 2021.

qui fait l'objet de l'article 13, ne couvre que les employeurs dans le domaine agricole. Cela étant, le Gouvernement est défavorable à ces dispositions comme il était défavorable à l'adoption de l'article 13 à l'Assemblée nationale. l'Assemblée nationale. Nous avons mis en place un système d'exonération de cotisations patronales et de crédits pour le paiement des cotisations salariales applicable à l'intégralité du secteur économique, sous réserve de pouvoir sous réserve de pouvoir démontrer une perte d'activité de 50 % pour les secteurs S1 et d'être fermé par décision administrative pour le secteur S1.

que nous nous interrogions sur la constitutionnalité de l'amendement qui a été adopté et qui est devenu l'article 13. Cet argument vaut également devant le Sénat. Enfin, autre difficulté pour la question des indépendants, des indépendants, dans un certain nombre de cas, l'adoption de l'amendement n° 428 rectifié proposé par Mme Delattre pourrait amener une prise en charge moins favorable pour les viticulteurs indépendants que ce que nous prévoyons dans le dispositif d'exonération déjà acté par le Gouvernement. Pour ce qui concerne les indépendants et uniquement eux, nous avons prévu, dans la mesure où la cotisation est annuelle, un dispositif d'exonération forfaitaire à hauteur de 600 euros par mois. prévu dans l'amendement n° 428 rectifié aux indépendants du secteur de la viticulture- je concentre mon propos sur celui-ci puisque j'ai entendu M. le rapporteur dire que la commission avait un tropisme favorable pour cet amendement

Voilà la différence négative pour les indépendants. La différence positive, mais j'ai exprimé ma crainte sur le caractère constitutionnel d'une telle mesure, serait pour les indépendants qui ne pourraient justifier d'une perte de chiffre d'affaires

Cela étant, et en nous en tenant aux arguments que nous avons développés en vain devant l'Assemblée nationale, nous considérons que la différence de traitement proposée au travers de ces amendements, comme d'ailleurs la différence de traitement intégrée dans l'article 13, ne se justifie pas entre les secteurs économiques. Le dispositif que nous avons prévu s'applique à l'ensemble des secteurs économiques sans risque juridique. Pour toutes ces raisons, le Gouvernement est défavorable à ces quatre amendements.

de chiffre d'affaires global dans l'ensemble de l'économie. Quand vous avez 30 % en moins, c'est un chiffre considérable : c'est tout un secteur qui s'effondre par pans entiers, surtout s'il est constitué par de petites exploitations, avec des surfaces minimes.

en termes de dispositifs de réduction des charges. C'est la raison pour laquelle je soutiendrai l'amendement de mon collègue Sebastien Pla, qui s'adresse à l'ensemble de ces filières. Si nous adoptions un dispositif ne concernant qu'une seule filière,

cette aide à partir de règles uniques pour tous les secteurs d'activité économique et de manière extrêmement limitée dans le temps. J'ajoute que la plupart des amendements- c'est une question de forme, mais cela peut compter -ne sont pas d'une totale clarté sur les périodes d'application

et sur la question des stocks en particulier, je rappelle à votre assemblée que nous avons d'ores et déjà rendu disponibles plus de 210 millions d'euros de crédits pour la distillation de crise, auxquels s'ajoute une quarantaine de millions d'euros pour aider les différents acteurs de la filière. Je pense notamment à ceux de la transformation.

de sauver des filières qui utilisent de la main-d'oeuvre locale dans nos départements de Guadeloupe et de Martinique. La filière canne-sucre-rhum nécessite que l'on prenne en compte à la fois les difficultés des entreprises, mais aussi

est à Mme Laurence Cohen. Selon l'Observatoire des multinationales, un tiers des entreprises du CAC 40 ont distribué des dividendes pendant la crise sanitaire, soit près de 30 milliards d'euros ainsi versés. Certes, c'est moitié moins qu'en 2019, où le montant atteignait 64,5 milliards d'euros, mais, contrairement à la crise sanitaire, la crise économique ne touche pas tout le monde de la même façon.

du chômage partiel pour 31 milliards d'euros, des reports ou annulations de cotisations sociales et de charges fiscales pour 76 milliards d'euros. Aider les entreprises en période de crise se justifie quand il s'agit des plus fragiles, mais pas de celles du CAC 40 qui profitent de la crise

ont bénéficié du filet de sécurité de notre sécurité sociale, il serait parfaitement logique de soumettre à cotisations sociales leurs revenus financiers. Face à l'urgence sanitaire et à la nécessité de trouver de nouvelles recettes pour financer notre système de santé, nous proposons donc de mettre à contribution les montants versés aux actionnaires aux taux actuels des cotisations sociales employeurs de la sécurité sociale. Il s'agit aussi d'une incitation forte pour les entreprises à privilégier le facteur travail. Mes chers collègues, ces nouvelles recettes sont importantes. Elles éviteraient

absolument scandaleux que le Gouvernement ne donne pas un signal aux gens qui en ont besoin.

soit grâce à la baisse des impôts de production, au chômage partiel, aux aides de la Banque centrale, aux plans sectoriels ou aux prêts garantis par l'État, 100

l'activité physique en milieu professionnel diminue de 32 % les arrêts de travail, soit une économie potentielle de 4,2 milliards d'euros par an. Elle diminue les troubles musculo-squelettiques et augmente la productivité de 12 %.

13 au PLFSS qui vient tout simplement effacer le dispositif adopté par les deux chambres : quel mépris à l'encontre du Parlement ! Après discussion avec l'ensemble des parties, nous avons travaillé à une nouvelle rédaction plus précise et, surtout, plus efficace

d'améliorer le texte. Nous étions, en effet, en désaccord sur la notion d'avantage sportif qui restait difficile à préciser en droit, sur la progressivité des aides accordées par les instances sociales des entreprises et sur le plafonnement éventuel de ce type d'avantage.

lorsque celui-ci se rattache à des activités sportives. Lors de l'examen à l'Assemblée nationale, le Gouvernement a supprimé cette mesure qui avait été introduite par un amendement sénatorial au projet de loi ASAP. Cette suppression est préjudiciable et constitue un frein supplémentaire au développement de la pratique du sport par les salariés.

applicable aux entreprises ultramarines, pendant une durée de deux années- du 1 janvier 2021 au 31 décembre 2022 -, qui correspond à la durée effective du plan de relance et du plan Logement outre-mer (PLOM).

Il serait préjudiciable à notre économie que ces entreprises disparaissent, licencient ou ne puissent pas embaucher les jeunes qui s'apprêtent à entrer sur le marché du travail.

ultramarines de BTP du régime de compétitivité renforcée pour le paiement des cotisations dues pour l'année 2021, afin de maintenir l'outil productif et de sauvegarder les emplois dans l'attente d'une reprise de l'activité, espérée pour 2022. La Merci,

À quel moment nous assoirons-nous raisonnablement autour d'une table pour comprendre que l'inactivité, dans ladite « outre-mer », coûte beaucoup plus cher que l'activité ? Lorsque nous demandons ces boîtes à outils pour régler au mieux les dispositifs, c'est parce que nous sommes conscients de

Cet amendement a pour objet de permettre aux établissements privés de santé d'être soumis au barème renforcé du régime d'exonération de charges sociales patronales spécifique applicable aux entreprises ultramarines, pour une durée de deux années- du 1 janvier 2021 2021 au 31 décembre 2022 -, dans une logique de différenciation, afin de tenir compte des difficultés spécifiques rencontrées par la filière réunionnaise depuis plusieurs années.

fortement créatrices d'emploi, ne peuvent pas toujours, paradoxalement, bénéficier du régime renforcé d'exonération de charges sociales patronales, alors que leur domaine d'activité

actuel, tant conjoncturel que structurel, cet effet de seuil, qui prive les entreprises de taille intermédiaire, dans les secteurs prioritaires, du bénéfice du principal régime d'aide en faveur de la compétitivité et de l'emploi, constitue un non-sens économique et social. social. Je vous demande donc de voter cet amendement pour que ces entreprises ne disparaissent pas de nos territoires.

Je suis désolé, je vais répéter les mêmes arguments ... On ne peut pas indéfiniment étendre un régime d'abattements très dérogatoire et assécher indéfiniment, de ce fait, les ressources de la sécurité sociale.

et, dans un élan de grande lucidité, vous déchirerez les arguments que vous venez de nous lire, vous verrez. Cela ne tient pas, monsieur le rapporteur général ! Faites-nous confiance, écoutez-nous, soyez à notre écoute

Cet amendement vise à rendre cohérents les différents dispositifs d'exonération de charges applicables dans les outre-mer avec les taux du régime dit « de compétitivité renforcée Ce régime représente le niveau intermédiaire d'exonération de charges entre celui, plus faible, dit « de compétitivité » et celui, plus fort, dit « innovation et croissance ». Le seuil de rémunération avant lequel les exonérations sont totales et à partir duquel elles deviennent dégressives a été porté, l'année dernière, en loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, à 2 SMIC pour le régime « de compétitivité renforcée ». Or ce même seuil, en régime « innovation et croissance », reste, lui, à 1,7 SMIC. dit, le régime d'exonération qui se veut le plus favorable ne l'est en fait pas pour les salaires compris entre 1,7 SMIC et 2 SMIC. Par cohérence, il convient donc de rehausser ce seuil pour le régime dit « innovation et croissance » et de le porter également à 2 SMIC. Quel est l'avis de la commission ? Alors qu'il existe

pour motif de sanctionner les dépassements d'honoraires abusifs. Malheureusement, elle s'applique aussi aux pédicures-podologues, dont les prestations ne sont pas prises en compte par l'assurance maladie ou le sont à des niveaux extrêmement faibles et qui se trouvent donc pénalisés par cette surcotisation qui,, ne devrait pas les viser. Il est donc proposé de mettre fin à cette situation qui est très mal ressentie par ces professionnels auxiliaires de santé.

est aussi une contrepartie à la participation financière de l'assurance maladie au paiement des cotisations sociales dues par ces praticiens au titre de leurs revenus conventionnés. Il nous semble donc qu'adopter ces dispositions irait contre ce système de régulation. La parole est à M. Arnaud Bazin,

que la formation continue obligatoire des professionnels de santé ou les activités qu'ils peuvent avoir au sein d'unions régionales de santé ou encore lorsqu'ils sont maîtres de stage ou en formation conventionnelle et syndicale. L'ensemble de ces professionnels sont aujourd'hui victimes d'un traitement inéquitable. La suppression de cette taxe irait dans le sens de ce que vous souhaitez, à savoir l'harmonisation des cotisations sur les revenus d'activité et un alignement des droits entre les professions.

Cette suppression est réclamée depuis longtemps par les syndicats et les départements, afin d'aider à financer la revalorisation de la prime de feu, sur laquelle il y a eu beaucoup d'engagements publics, comme chacun le sait ici. L'annulation de cette surcotisation permettrait, en effet, de dégager une enveloppe de 40 millions à 45 millions d'euros pour les employeurs et, ainsi, d'aider à financer la revalorisation de la prime de feu de 19 % à 25 %.

il a simplement accepté de supprimer la part employeur dont s'acquittent les SDIS, c'est-à-dire essentiellement les départements, avec pour objectif d'améliorer les finances départementales et d'augmenter le pouvoir d'achat des sapeurs-pompiers professionnels.

Il est vrai que le budget des services départementaux d'incendie et de secours pèse de plus en plus sur les conseils départementaux et que les concours de l'État sont urgents et nécessaires. Cela n'est pas mis en cause, cause, mais, pour des raisons de cohérence, d'équité et de justice, notre amendement tend à supprimer également la part salariale de la surcotisation, actant ainsi la suppression totale de celle-ci, qui, d'ailleurs, aurait dû

vise aussi à supprimer la surcotisation salariale. Je partage ce qui vient d'être dit sur le fait que le Gouvernement n'est pas allé au bout- l'Assemblée nationale non plus, du reste. Je rappelle à mon tour que cette surcotisation a été instituée en 1990 pour financer l'intégration progressive de la prime de feu dans les pensions de retraite des sapeurs-pompiers. Alors qu'elle avait vocation à s'éteindre en 2003, elle a perduré jusqu'à aujourd'hui. L'intégration de la prime de feu est désormais effective, le nombre de cotisants a progressé de 10 000 et le nombre de ceux qui partent à la retraite sans avoir cotisé au titre de cette prime de feu diminue : il n'y a donc pas de problème proprement financier, me semble-t-il. Aujourd'hui, le Gouvernement, après de très fortes mobilisations des sapeurs-pompiers, a décidé de revaloriser la prime de feu, ce qui est une très bonne chose. La suppression de

Le décret a été signé par le ministre de l'intérieur. Le relèvement du plafond de 19 % à 25 % permet une augmentation de la rémunération nette de 100 euros. Dans la discussion Dans la discussion avec l'Assemblée des départements de France, la question du financement de cette augmentation a été posée. Le Gouvernement, par la voix du ministre de l'intérieur, s'est engagé à supprimer la surcotisation patronale, ce que nous avons fait à l'Assemblée nationale,

que l'engagement d'augmenter la prime de feu a été tenu, que la suppression de la surcotisation patronale est un élément de financement de cette augmentation, qui est à la charge des SDIS, et que la suppression de la surcotisation salariale ne nous paraît pas opportune, compte tenu de sa dimension contributive.

: vous avez affirmé, madame la sénatrice, que le Gouvernement aurait cédé à la mobilisation des sapeurs-pompiers. Je peux vous assurer que cette mobilisation était légitime et que la demande d'augmentation de la prime de feu- je ne parle pas du dispositif d'exonération

et souvent intéressante dans les zones de désertification médicale. Ces centres sont des lieux de santé de proximité qui assurent des activités de soins sans hébergement et participent à des actions de santé publique, de prévention et d'éducation pour la santé. Une approche globale de la santé est favorisée autour des médecins, de l'ensemble des professionnels médicaux et paramédicaux, des patients et des citoyens. La gestion administrative est mutualisée. À l'heure actuelle, ces centres sont gérés sous la forme associative ou relèvent des collectivités locales. Pourtant, en 2016, la loi de modernisation de notre système de santé a permis la création de centres de santé sous la forme de sociétés coopératives d'intérêt collectif (SCIC). Cette possibilité a ensuite été précisée par l'ordonnance du 12 janvier 2018. La gouvernance multipartite du statut coopératif permet d'associer les professionnels de santé, le personnel les patients à la gestion, instaurant ainsi une démocratie sanitaire locale tout à fait intéressante. Dans la réalité, il est nécessaire de compléter le cadre législatif en adoptant des dispositifs fiscaux assurant l'équilibre financier de ces entreprises coopératives non non lucratives. Nous proposons donc d'aligner leur cadre fiscal sur celui des associations gérant ces mêmes centres. En effet, sous statut coopératif, les centres de santé permettent le bénéfice de la décote pour la taxe sur les salaires dont bénéficient les associations, soit, en 2020, un montant de 21 044 euros par établissement. Cet amendement vise donc à instaurer deux dispositions qui permettront aux centres de santés établis sous statut de SCIC d'atteindre leur équilibre financier,

coopérative d'intérêt collectif constitue une forme sociale commerciale spécifique. C'est l'ordonnance du 12 janvier 2018 relative aux conditions de création et de fonctionnement des centres de santé qui a permis à ces derniers de se constituer sous la forme de SCIC. Ces centres de santé, comme tous les acteurs du secteur hospitalier et médico-social, sont soumis à la taxe sur les salaires. Compte tenu de leur forme juridique, ils ne peuvent bénéficier de l'abattement de cotisations de 21 044 euros auquel sont éligibles les associations relevant

Une telle extension à des structures constituées sous une forme commerciale, certes particulière, fragiliserait le mécanisme au regard du principe d'égalité devant les charges publiques et pourrait créer des distorsions de concurrence vis-à-vis d'employeurs qui n'ont pas cette forme juridique, mais qui réalisent des activités identiques et dans des conditions comparables, comme les établissements de santé publics ou privés. Les exonérations en matière fiscale doivent, selon nous, viser des objectifs spécifiques sans porter atteinte

Cet allégement représente une perte de recettes annuelle de 22 milliards d'euros pour l'assurance maladie. Compensé en partie, il est accordé aux entreprises sans contrepartie.

un soubassement idéologique, celui du coût du seul facteur travail, et un point aveugle, celui du coût du capital, notamment du capital

La Cour de justice de l'Union européenne a considéré que cette imposition n'était pas conforme au droit européen.

Pour autant, les non-résidents continuent d'être assujettis à l'imposition à hauteur de 17,2 % et paient également, dans les pays de résidence,

Ce n'est pas une bonne chose : un tel dispositif aurait pour effet d'exonérer de CSG et de CRDS les revenus immobiliers de tous les non-résidents, y compris ceux qui relèvent d'un régime obligatoire de sécurité sociale français. Concrètement, cela reviendrait à exonérer les personnes qui ont effectué toute leur carrière professionnelle en France et qui s'expatrient en Espagne ou au Maroc, par exemple, au moment de leur retraite. La solution de M. Cadic n'est pas non plus satisfaisante, puisqu'il propose non seulement d'exonérer de CSG et de CRDS les non-résidents qui sont à la charge d'un régime obligatoire de sécurité sociale français, mais aussi de remettre en cause l'application de la jurisprudence dite et d'assujettir de nouveau à la CSG des résidents qui relèvent du régime obligatoire de sécurité sociale d'un pays de l'Union européenne.

sans distinction géographique. Cela fait six ans que nous défendons cette idée chaque année dans l'hémicycle. La Cour de justice de l'Union européenne a d'ailleurs jugé cette disposition contraire au droit européen. La loi du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 a abrogé ces cotisations pour les seuls résidents de l'Union européenne, de l'Espace économique européen et de la Suisse. Cette fiscalité à deux vitesses est vécue comme une terrible injustice par les Français de l'étranger demeurant assujettis. Surtout, elle est constitutive d'une discrimination violant le principe constitutionnel d'égalité devant la loi fiscale. la loi fiscale. Cet amendement du sénateur Cadic vise donc à mettre le droit positif en cohérence avec nos principes constitutionnels en exonérant de prélèvements sociaux- CSG, CRDS et autres -sur les revenus du patrimoine de source française l'ensemble des 3,5 millions de Français non résidents non affiliés à un régime français

s'agit d'un amendement déposé par notre collègue Jean-Yves Leconte. Le Gouvernement a proposé dans le PLFSS pour 2019 la suppression de l'assujettissement à la CSG et à la CRDS des revenus du capital des personnes non résidentes fiscales, mais installées dans l'Espace économique européen et en Suisse. En effet, le principe d'unicité de la législation applicable posé par l'article 11 du règlement n° 883/2004 engendrait pour l'État un risque contentieux important si les dispositions existantes n'étaient pas modifiées. Toutefois, la subsistance d'un impôt visant exclusivement certains non-résidents et non d'autres en fonction de leur lieu de résidence heurte le principe constitutionnel d'égalité devant l'impôt. Il est donc proposé d'étendre la suppression de l'assujettissement à à l'ensemble des non-résidents non assujettis à un régime de protection sociale français, comme le réclament nombre de Français non installés dans l'Espace économique européen ou en Suisse et devant faire face à ce prélèvement injuste. Rappelons enfin que cet amendement a été voté en première lecture au Sénat comme article 21 de la proposition de loi relative aux Français établis hors de France présentée par le sénateur Retailleau. Il est donc cohérent que cet amendement soit aussi voté dans le cadre de ce PLFSS.

Or les Français résidant hors de France ne bénéficient ni de la sécurité sociale, ni de l'école gratuite, ni de l'assurance chômage, ni des allocations familiales, ni de la retraite. En revanche, ils payent des impôts sur leurs salaires, retraites et pensions d'origine française, ce qui est normal. Ils paient également des impôts sur leurs revenus immobiliers, c'est-à-dire sur l'appartement qu'ils ont en France et qu'ils ont loué pour rembourser leur crédit en attendant qu'il puisse leur servir à payer leur retraite. Ils payent donc un impôt de 30 % sur leurs revenus français, ce qui, encore une fois,

réduit de moitié. Les Français résidant à l'étranger dans l'Union européenne, en Suisse et dans l'Espace économique européen ont dû aller devant la Cour de justice de l'Union européenne pour obtenir d'être exonérés de CSG-CRDS. Mais les Français de l'étranger résidant hors de l'Union européenne, de la Suisse et de l'Espace économique européen ne sont toujours pas C'est une injustice flagrante, une situation totalement discriminatoire. Je compte donc sur vous tous, mes chers collègues, pour nous aider à réparer cette injustice et voter la suppression de la CSG-CRDS sur les revenus mobiliers de tous les Français résidant hors de France.

négociation de règles relatives aux doubles impositions, comme cela a été fait avec les États-Unis, ou par le renoncement de la France à une partie de sa fiscalité, qui coûterait 300 millions

Je vous le rappelle, en 2014, le Conseil d'État a rendu un arrêt relatif à une vente d'immeuble en SCI par des non-résidents d'un pays tiers à l'Union européenne, qui devaient s'acquitter des prélèvements libératoires de 33,33 %. Les non-résidents européens ayant à payer un taux inférieur à celui des pays tiers, le Conseil d'État a estimé que cette différence de traitement constituait une restriction aux mouvements de capitaux. Il semble donc que le sujet puisse encore, monsieur le ministre, évoluer.

Nous les avons votés dans le cadre d'une proposition de loi. Je considère qu'il y a une discrimination en fonction de la géographie et que nos

de la valeur ajoutée par l'entreprise. Je pense, d'une part, à l'intéressement et, d'autre part, à la participation aux résultats de l'entreprise. On constate que, dans les entreprises de petite taille - les PME de moins de 250 salariés et, singulièrement, les entreprises de moins de 50 salariés -ces dispositions sont encore très peu usitées. Or on voit bien qu'il serait conforme à l'intérêt général que le pouvoir d'achat des uns et des autres soit amélioré, et ces outils sont des vecteurs intéressants pour agir en ce sens. Ainsi, pour encourager le recours à ces dispositifs, je propose de supprimer le forfait social pour les entreprises de moins de 250 salariés s'agissant de la participation aux fruits de l'expansion de l'entreprise et de l'intéressement.

pour favoriser la participation et l'intéressement : nous avons simplifié les procédures et diminué le forfait social et les prélèvements qui pèsent sur ces sommes. Nous considérons avoir atteint un niveau d'incitation

dispositifs dont bénéficient les salariés. S'ils ne peuvent pas avoir de retraite chapeau, il est indispensable qu'ils bénéficient d'une amélioration de leur pouvoir d'achat, et en particulier qu'ils puissent recueillir les fruits de l'expansion de l'entreprise. Or, aujourd'hui, les versements de l'entreprise sont taxés à 20

J'entends bien les arguments de Michel Canevet. Si j'ai bien compris, l'amendement vise à faire passer le taux du forfait social de 20 % à 10 %. %. L'alignement sur le taux de l'abondement en actionnariat salarié ne paraît pas souhaitable, mettant sur le même plan l'amplification d'un effort du salarié et un complément de rémunération versé sur la seule initiative de l'entreprise. Je ne suis pas sûr que ce soit exactement ce que recherche Michel Canevet.

à Mme Laurence Cohen. Le Gouvernement a transformé le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi en suppression définitive des cotisations des entreprises à la branche famille de la sécurité sociale. Cette décision a entraîné la perte de 20 milliards d'euros de cotisations, la remise

Alors que le CICE a coûté près de 125 milliards d'euros, il serait temps de s'interroger sur l'utilité de ces exonérations de cotisations sociales pour l'emploi. En décembre 2018, l'Insee a estimé que la bascule

150 000 emplois supplémentaires pour 60 milliards d'euros en 2021. Cela représente tout de même 400 000 euros pour la création d'un seul emploi Le Conseil d'analyse économique avait d'ailleurs été bien plus sévère sur l'effet de la transformation du CICE. Permettez-moi de le citer : « Le gain pour les entreprises est nul, car seule change la forme. » Pour toutes ces raisons, nous proposons de rétablir les cotisations patronales à la branche famille,